mes chers collègues, que la conférence des présidents a prévu que nous siégions ce matin et cet après-midi jusqu'à

et aux ministres, personne ne comprendrait que le candidat à la présidence de la République ne les donnât point. En se focalisant sur le patrimoine du Président de la République, la loi de 1962, déjà ancienne, fait l'impasse sur la deuxième partie de l'article LO 135-1 du code électoral auquel il se réfère, alors que la campagne présidentielle a démontré la pertinence qu'il y aurait à exiger une déclaration d'intérêts aux candidats à cette élection. Il ne vous aura pas

représente, selon nous, une atteinte caractérisée à la démocratie. Ainsi, les médias et les instituts de sondage seraient légitimes à décider quel candidat est digne de s'adresser aux Françaises et aux Français. Pour ce faire, ils s'appuieraient, d'une part, sur la « capacité d'animation » des candidats- expression le potentiel de « buzz » et de polémiques -, et, d'autre part, sur les résultats antérieurs desdits candidats. Ces deux éléments entraînent trois conséquences majeures. Premièrement, ils empêchent l'émergence de nouvelles forces, puisque des résultats antérieurs conditionnent l'exposition. Deuxièmement, ils encouragent la perpétuation de scrutin en scrutin des mêmes rapports de force. En effet, une formation ayant obtenu de bons résultats serait plus exposée et aurait donc plus de chance de maintenir son niveau de vote. Troisièmement, ils transforment le débat de fond

Cet amendement vise donc à revenir sur la réforme de 2016 en réinstaurant l'égalité du temps de parole pour l'ensemble de la campagne, et ce dès la parution du décret de convocation des électeurs. Ainsi seront concernés les candidats à l'élection présidentielle dans leur ensemble, mais aussi les candidats putatifs à la recherche de leurs parrainages d'élus. Nous considérons

dernière élection présidentielle a montré que même cette loi scélérate- disons-le !-n'a pas été respectée. On a eu affaire à un festival d'inégalités et de n'importe quoi comme on n'en a jamais vu

Il s'agit de réduire de moitié les plafonds de dépenses pour les campagnes électorales en vue de l'élection présidentielle, en passant de 13,7 millions à 6,85 millions d'euros pour tous les candidats à l'élection, et de 18,3 millions à 9,15 millions d'euros pour les deux candidats encore en lice au second tour. malgré des efforts de contrôle et de transparence depuis trois décennies, les scandales se sont multipliés. Entre les meetings, les déplacements et l'impression des tracts, les dépenses de certains candidats peuvent atteindre des sommets. Pour éviter des abus et de possibles dérapages, des règles et un encadrement du financement des campagnes électorales ont été mises en place depuis la fin des années quatre-vingt. Mais force est de constater, à la suite de la dernière campagne en vue de l'élection présidentielle, que les choses pourraient être davantage clarifiées et encadrées. Pour assainir quelque peu ces dépenses, et les moraliser, nous proposons de les diminuer. Dans un souci de bonne utilisation des deniers publics, ces sommes faramineuses ne se justifient pas,

L'argent pollue la sphère publique, et plus encore à l'ère de la communication excessive et des campagnes tape-à-l'oeil. Aux candidats à la plus haute fonction de l'État de montrer l'exemple en se satisfaisant de campagnes moins onéreuses à tous les niveaux, lesquelles feront davantage appel à l'intelligence des électeurs et à l'intérêt pour le débat public.

zéro ». Après tout, la possibilité de s'exprimer à la télévision devrait suffire ! Or il se trouve que les campagnes présidentielles mobilisent tout de même nombre de nos concitoyens,

du Gouvernement ? Madame la sénatrice, le Gouvernement ne vous suivra pas dans votre proposition. Nous considérons en effet que l'objet de la loi est non pas de diminuer le montant des dépenses électorales, mais d'assurer leur transparence, ce qui est une première raison de refuser cet amendement. J'ajoute que le montant des dépenses électorales n'a pas été réévalué depuis 2009, ce qui conduit, de fait, à une diminution du plafond des dépenses.

est à Mme la garde des sceaux. Compte tenu de la possibilité offerte aux élus en retard de déclaration et de paiement de se mettre en conformité avec leurs obligations fiscales, sur invitation expresse de l'administration fiscale, il ne nous semble pas justifié, en cas de manquement persistant à cette obligation, de réduire le champ d'application de la démission d'office aux seuls manquements caractérisés par une particulière gravité. Il nous semble également qu'il n'y a pas lieu de donner au bureau de chaque assemblée un pouvoir d'appréciation du manquement. Je rappelle, au demeurant, que la suppression du critère de particulière gravité n'empêchera pas le Conseil constitutionnel d'exercer un contrôle de proportionnalité de la sanction en tant que juge de l'élection. Cela me conduit donc, je le dis d'ores et déjà, à être favorable au sous-amendement qui a été déposé

n'est pas en règle avec ses obligations fiscales les plus élémentaires, la transmission au bureau de l'assemblée, lequel n'est pas une simple boîte aux lettres, se fait

du manquement. J'admets, madame la garde des sceaux, comme nous l'avons fait pour les parlementaires européens, qu'il ne faille pas poser l'exigence d'un manquement d'une particulière gravité, mais permettre au Conseil constitutionnel d'avoir une appréciation en fonction de la gravité du manquement. C'est subtil,

Cet amendement vise à imposer aux candidats à l'élection présidentielle ou aux élections législatives et sénatoriales la production d'un casier judiciaire vierge. Je ne reviendrai pas sur les arguments que j'ai développés lors de la

Par ailleurs, en ce qui concerne la comparaison que vous avez faite avec l'accès à la fonction publique, il me semble que le droit de suffrage a un caractère constitutionnel extrêmement puissant,

et pose comme règle que les maires de communes de plus de 3 500 habitants ne peuvent pas faire plus de trois mandats. Je sais bien que votre intention est de protéger les maires des communes de moins de 3 500 habitants. Mais êtes-vous sûr d'être réellement favorable à à la limitation de la souveraineté de l'électeur, qui se verrait interdire de renouveler pour un quatrième mandat le maire d'une commune de 3 502 habitants

est un droit fondamental. Si nous adoptions une disposition, comme le Gouvernement l'avait souhaité, qui limite dans le temps le renouvellement des mandats, il faut réviser la Constitution. C'est si vrai

de la nature juridique du lien entre ces personnes et leur employeur, qui, lui, est public et exerce des responsabilités

d'empêcher d'être candidats des personnalités qui pourraient, par les responsabilités qu'elles exercent,

Marie-France Beaufils. Des élus sont régulièrement sollicités par des concitoyens, des associations et aussi des groupes d'intérêts. Ces sollicitations peuvent s'accompagner d'un cadeau, d'une invitation, voire d'une ristourne au montant parfois élevé. Certains groupes d'intérêts espèrent obtenir compensation de ces cadeaux. Dans l'esprit de ce qui nous a animés lors des dernières années où plusieurs réformes ont vu le jour, comme la déclaration de patrimoine et le registre des représentants d'intérêts, il s'agit aujourd'hui pour nous d'aller plus avant dans la prévention des conflits d'intérêts et de lever les soupçons réguliers de corruption. Les récentes échéances Les récentes échéances électorales ont marqué l'attention particulière des Français au sujet des cadeaux faits aux élus. Cette exigence de transparence traduit la perte de confiance des citoyens envers leurs élus, qu'il nous convient de restaurer, en inscrivant dans le projet de loi organique dont nous débattons un principe de prudence. Ainsi, nous proposons d'ajouter l'obligation de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la nature, la valeur, l'origine et le motif de tout avantage gratuit excédant une valeur de 1 500 euros.

Nous avons adopté des règles depuis mai 2015. Cette obligation est assortie de sanctions disciplinaires.

Il ne s'agit évidemment pas d'empêcher les personnes assurant ces fonctions de devenir parlementaires : leur expérience dans l'entreprise peut utilement éclairer le débat public. Il est cependant nécessaire de les contraindre de choisir entre la faculté d'exercer ponctuellement un mandat de représentant de la Nation et des engagements professionnels potentiellement très lourds. Le mandat parlementaire exige une très grande disponibilité, on l'a régulièrement entendu dans le débat sur le non-cumul des mandats. La direction d'entreprises de plus de 5 000 salariés ou générant un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards d'euros, avec

Ma chère collègue, la nature du problème est exactement la même, que la société soit petite ou grosse. Les incompatibilités sont faites pour éviter que les liens d'intérêts d'un parlementaire mettent en cause son indépendance. Vous savez que les incompatibilités sont, heureusement, déjà très larges puisqu'elles comprennent le fait de travailler pour des sociétés cotées, des sociétés d'économie mixte, des sociétés subventionnées par la puissance publique. Mais que la société soit petite ou grosse, rien du point de vue de la protection de l'indépendance du parlementaire. C'est la raison pour laquelle je vous serais très reconnaissant si vous acceptiez de retirer votre amendement au bénéfice des explications que je vous ai apportées.

Le projet de loi organique prévoit que les parlementaires qui exercent une activité de conseil sont autorisés à poursuivre une telle activité si celle-ci a été initiée dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction. Notre volonté est de faire que cette loi soit efficace et qu'elle garantisse une confiance totale de nos concitoyens dans l'action publique, sans pour autant sombrer, comme cela a été rappelé plusieurs fois, notamment lors de la discussion générale, dans une chasse aux sorcières qui serait néfaste. Le présent amendement prévoit que le parlementaire est autorisé à poursuivre une activité de conseil si celle-ci a été initiée dans les trois ans précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction. Cet amendement vise à lever tout soupçon à l'encontre des parlementaires concernés. En effet, le délai de douze mois, initialement prévu, ne nous semble pas suffisant pour garantir la plus grande transparence vis-à-vis de nos concitoyens. Vous le savez, douze mois avant l'élection, dans de nombreux cas nous connaissons déjà les candidats qui se présenteront. Il s'agit de prévenir les situations dans lesquelles certains d'entre eux tenteraient de développer une activité de conseil en vue de devenir parlementaire. C'est pourquoi le délai proposé nous semble insuffisant. Sans sombrer dans une suspicion systématique, nous ne devons pas laisser de place aux doutes pour nos concitoyens et nous devons faire preuve de la plus totale transparence. Quel

mesure est gravement frustratoire d'un droit fondamental : celui de tout Français d'être candidat à une élection. Je pense même que, en ayant prévu un délai d'un an

Mme Éliane Assassi. À défaut d'interdire l'activité de conseil aux parlementaires en cours de mandat, nous souhaitons, au travers de cet amendement, limiter les revenus annexes tirés de ces activités.

Il s'agit, même si l'activité de conseil du parlementaire est en sommeil, de permettre une traçabilité des possibles conflits d'intérêts. Au travers d'une contribution du groupe CRC à une mission d'information sur les conflits d'intérêts, menée par l'ancien sénateur Jean-Jacques Hyest, nous étions même allés plus loin

activité. Par ailleurs, nous préconisons d'aller beaucoup plus loin dans le régime des incompatibilités, en interdisant notamment tout travail pendant l'exercice d'un mandat. Le caractère général de cette interdiction aurait au moins le mérite de la clarté.

de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, cet amendement tend simplement, à défaut de l'interdire, à limiter la proportion des revenus issus des activités de conseil. Il s'agit donc d'un amendement de repli et, me semble-t-il, de bon sens.

c'est quelque chose d'un peu surprenant pour la grande majorité de nos concitoyens, mais c'est le droit -et, d'autre part, l'exigence d'indépendance ainsi que celle de disponibilité.

notre raisonnement consiste à dire que, quand l'activité professionnelle de conseil prend un caractère prédominant par rapport à l'exercice du mandat parlementaire, si l'on ne peut constitutionnellement s'y opposer- c'est d'ailleurs pour cela que les amendements consistant à plafonner légalement les ressources

que l'intéressé, qui perçoit donc plus de 150 000 euros par an de son activité de conseil, indique dans sa déclaration d'intérêts qui sont les cinq premiers contributeurs.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a des activités qui, avec trois ou quatre heures de travail, peuvent apporter une rémunération

en prévoyant que l'on ne peut conserver une activité de conseil qui n'aurait pas été commencée au moins un an

par le secret professionnel. Cela dit, je dois dire que l'entorse à nos principes que constituerait cette disposition me paraît infiniment moins grave

l'indemnité parlementaire, n'établit pas une interdiction absolue, mais, malgré cela, le fait de limiter les revenus tirés d'une activité, quelle qu'elle soit, est susceptible de porter atteinte à la liberté d'entreprendre. En outre, l'objectif visé, tout à fait digne d'intérêt puisqu'il s'agit d'inciter fortement les parlementaires à se consacrer à l'exercice de leur mission et à leur mandat,

Merci

Le scrutin est ouvert.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

Bien que je souhaite permettre aux représentants de la Nation de travailler, cela doit évidemment être encadré et soumis à certaines règles. C'est pourquoi je propose que les revenus tirés des activités de conseil soient plafonnés à un seuil de 50 % de l'indemnité parlementaire, limiterait ainsi le risque de conflit d'intérêts sans engendrer de suspension ou de cessation forcée d'activité. En effet, je le rappelle, la politique n'est pas un métier, mais bien un mandat, une fonction ; elle ne doit donc être que momentanée.

non pas d'inciter les parlementaires à se consacrer à leurs affaires personnelles plutôt qu'à celles de la Nation, mais de leur permettre de conserver leur activité de conseil qui serait bien antérieure à leur prise de fonction d'élu du peuple, sans les pénaliser, le délai d'un an écartant ceux qui auraient anticipé ou souhaité un cumul des deux pour diverses raisons,

il est indexé sur le montant de l'indemnité parlementaire. Si vous considérez qu'il est préférable que cette obligation déclarative, qui n'empêche nullement l'activité,

pour une activité de conseil, choisit comme prestataire un parlementaire, dont toutes les activités politiques sont publiques, on peut considérer qu'il renonce

que certaines de ses décisions soient influencées par la part que prennent, dans ses activités et revenus, des clients spécifiques, raison pour laquelle on a précisément inventé les déclarations d'intérêts.

est par nature consubstantielle à la démocratie et que l'indépendance nécessaire pour être source d'information ne peut être compatible avec le fait d'exercer des fonctions de représentation politique.

aurait également pour effet de restreindre le droit de propriété des parlementaires, qui pourraient investir dans un certain nombre d'entreprises, mais pas dans des entreprises de presse, au motif que la presse, si je comprends bien, ne doit jamais exprimer d'opinion et doit se borner à relater des faits

au contraire la reconnaissance, dans la tradition républicaine, d'un engagement des parlementaires dans des activités de presse et de l'existence d'une presse d'opinion qui s'assume

protègent le parlementaire contre le risque de dépendre d'intérêts. Aucune incompatibilité ne peut être justifiée par d'autres motifs. Or la participation à une entreprise de presse,

ces amendements se heurtent à des principes fondamentaux, qui ne sont pas de pure forme et touchent à la liberté

a estimé devoir s'opposer à ces amendements. J'ajoute que j'ai été saisi par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, qui est toujours extrêmement sourcilleuse

pour les parlementaires qui siègent actuellement dans les conseils d'administration de Radio France ou de France Télévisions, de se retirer. C'est aussi un élément que nous devons prendre en considération. Souvent, j'entends des plaintes

mais on pratique souvent avec eux ce qui ressemble un peu à du trafic de reliques. Il est vrai que l'on ne manque pas de parlementaires qui furent aussi

décide de mettre en place une campagne de communication, sous couvert de publicité institutionnelle- avec argent sonnant et trébuchant

La commission des lois, sur avis de son rapporteur, Hugues Portelli, a estimé alors que ce procédé constituait une atteinte à la séparation des pouvoirs, le parlementaire devant se consacrer parallèlement à sa mission législative, de contrôle et d'évaluation au sein du Parlement.

permet au suppléant du député élu sénateur de siéger à sa place jusqu'au prochain renouvellement de l'Assemblée nationale. Cependant, lorsque ces deux élections se succèdent à quelques semaines d'intervalle, un député récemment élu faisant le choix d'être également candidat aux sénatoriales transmettra automatiquement, est élu, son siège de député à son suppléant, sans nouvelle élection. On voit ici parfaitement la manoeuvre consistant à mettre en avant un candidat à la forte notoriété pour gagner la circonscription et ensuite permettre au suppléant, moins connu, d'exercer le mandat quelques semaines plus tard, plus tard, sans permettre aux électeurs de valider cette succession. Le retour naturel aux électeurs nous paraît essentiel lorsque ce cas de figure se présente afin de permettre aux citoyens de choisir légitiment le député qu'ils souhaitent voir représenter

Louis Masson, pour explication de vote.

amendement prévoit que la désignation d'un parlementaire dans un organisme extraparlementaire ne peut se faire qu'en vertu d'une loi et non pas d'un décret.

se retrouver sans emploi ou condamné à faire un travail autre que celui pour lequel il est qualifié ? Pourquoi un ancien plombier ou un ancien cadre d'entreprise pourraient-ils retrouver du travail dans une entreprise,

d'anciens parlementaires issus du secteur public, auxquels on interdirait, puisqu'ils auraient rompu tout lien avec la fonction publique, de reprendre un travail de fonctionnaire ? Ce serait une injustice qui ne réparerait pas l'injustice dont sont victimes les anciens parlementaires

et une plus grande transparence. À cet égard, le dispositif actuel, à savoir la mise en disponibilité pendant l'exercice du mandat et le respect d'un certain nombre d'obligations déontologiques

est mon cas. Par ailleurs, ayant été élu relativement jeune, je suis assez sensible à ce que j'entends. La seule garantie que nous ayons, en entrant au Parlement, c'est l'obligation pour l'entreprise de nous mettre en suspension du contrat de travail, suspension valable une seule fois.

ce que nous recherchons

nous souhaitons tous que le Parlement soit la représentation la plus large de la réalité de notre société ; d'un autre côté, nous sommes en train d'accumuler obstacles et interdits à cette diversité. Selon moi, la compétence,

en métier politique de gens n'ayant jamais exercé aucun métier et qui ne se trouvent là où ils sont que par la grâce d'appareils politiques.

Tasca. Nous connaissons tous, aussi bien à gauche qu'à droite ou au centre, des personnalités entrées très jeunes dans la fonction publique, ayant ensuite exercé plusieurs mandats parlementaires

sur l'article. Le présent article visait initialement à supprimer purement et simplement la réserve parlementaire En jetant ce pavé dans la mare, le Président de la République et de son gouvernement ont fait le choix d'envoyer des signaux clairs : sous couvert de moraliser la vie politique, ils ciblent particulièrement les parlementaires et souhaitent limiter leurs financements et leurs prérogatives. Les parlementaires coûtent toujours trop cher et il faut limiter la dépense publique. Nous connaissons le laïus. Les travers antiparlementaristes de cette loi ne nous ont donc pas échappé. Pour autant, il s'agit d'une vraie question, tant la suspicion est forte, résultat des dérives constatées dans certains territoires. L'exigence de transparence d'aujourd'hui doit être prise en compte par les élus que nous sommes. En commission, cet article a été totalement réécrit pour concilier à la fois le maintien de la réserve parlementaire, tout en encadrant plus fortement son usage. Nous prenons connaissance pour la séance de trois séries d'amendements : certains parlementaires ne veulent finalement aucune contrainte sur l'usage de la réserve

la suppression de la réserve parlementaire signifie la limitation des ressources des territoires et des collectivités, sans oublier les associations durement frappées par l'austérité, nous ne sommes pas d'accord.

lors de la loi de finances, quels seront les arbitrages et nous vous rappellerons vos promesses. Ces 140 millions doivent rester au service des territoires et de leurs habitants. Pour nous, le débat doit essentiellement porter sur la question suivante : l'idée même d'une réserve parlementaire est-elle légitime ? En la matière, les avis sont partagés.

dont le délégué général était son assistant parlementaire, et dont la trésorière était sa première adjointe ! C'est quand même incroyable ! Pour couronner le tout, le siège de l'association se trouvait dans son bureau au Sénat ! Il y a quand même des limites ! Et les communes n'ont pas à être les victimes

la réserve parlementaire était distribuée dans une certaine opacité. Je me souviens qu'à mon arrivée dans cette maison,

votions des dispositions pour réformer cette immoralité. Mais aujourd'hui, grâce au travail effectué, la réserve parlementaire est totalement transparente. Il s'agit de sommes affectées à des communes,

C'est pourquoi nous considérons que ce sujet ne devrait pas intervenir dans le cadre de ce texte. Mais au cas, probable, où notre amendement ne serait pas adopté, nous nous rallierons à celui de la commission, c'est-à-dire au texte tel qu'il nous est présenté.

des dossiers dans chaque ministère, que ce soit à l'intérieur, surtout, ou aux affaires étrangères, à la culture, à la jeunesse et aux sports, aux affaires sociales.

attirer l'attention sur le fait suivant : cette dotation est menacée depuis très longtemps. Dès lors qu'il faut faire des économies, on gratte partout !

la réserve soit détournée de sa fonction pour financer des associations dont l'objet était tout à fait sujet à caution et dont les pratiques l'étaient encore